la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

peut l'être pour d'autres ! Et quand on a de l'ambition pour ce département d'Alsace, comment ne pas en avoir pour les autres départements ?

Tous les départements de France peuvent revendiquer des spécificités, qui justifieraient de leur confier des compétences exorbitantes du droit commun. Les départements du Nord, des Alpes-Maritimes, de Meurthe-et-Moselle, du Doubs, des Pyrénées-Orientales ou des Pyrénées-Atlantiques, ou encore leurs régions respectives, sont également des territoires frontaliers et devraient aussi pouvoir bénéficier des compétences accordées à l'Alsace. Les départements bretons, savoyards ou vendéens, ayant une identité culturelle au moins aussi affirmée que celle de l'Alsace, devaient aussi pouvoir bénéficier des compétences qui lui sont accordées. Aussi, afin d'éviter à ce projet de loi une potentielle censure partielle par le Conseil constitutionnel et en vertu des principes d'égalité et d'indivisibilité de la République, il est proposé de rétablir l'égalité en étendant à tous les départements les compétences confiées au futur département d'Alsace.

de l'Alsace comme région de plein exercice et la réduction de la taille de la région Grand Est. Vous comprendrez donc que nous essayions de compenser

se voient attribuer les compétences et prérogatives reconnues par l'article 1 au département d'Alsace. Nous y sommes favorables, car il n'y a aucune raison de de priver de ces attributions d'autres départements qui présenteraient des caractéristiques analogues à celles de l'Alsace. Très bien ! Je demande néanmoins deux légères rectifications : remplacer les mots « l'ensemble des compétences » par les mots « tout ou partie des compétences », parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de sens à attribuer à la Sarthe ou à la Drôme un chef de filât en matière transfrontalière

J'ajoute que le Gouvernement est tout à fait prêt à discuter avec les collectivités frontalières de toute politique transfrontalière adaptée à leur territoire. Je le dis haut et fort, et vous pouvez le transmettre à vos collectivités territoriales respectives. Mais, quand on veut faire, comme c'est l'objectif du Gouvernement, du « cousu main

des spécificités de l'Alsace, à ce point faibles qu'elles intéressent tous les départements de France et d'outre-mer. C'est très intéressant. On nous a dit que ce texte se fondait sur les spécificités de l'Alsace ; je note qu'il intéresse tout le monde,

Nous souhaitons appliquer les règles classiques, traditionnelles, par lesquelles notre pays a toujours réussi à concilier l'unité nationale avec la diversité locale. Cela suppose, pour y parvenir- et on peut très bien y parvenir que l'on revienne sur un ensemble de lois stupides qui ont détruit un ensemble institutionnel qui fonctionnait. Pour ce faire, il faut revoir dans le détail,

alors- je le pense -, selon notre logique, à concilier cette unité nationale avec les spécificités locales, comme on l'a toujours fait. Voilà ce que nous souhaitons.

du Cantal ! Voyez-vous, je n'ai pas attendu ce soir pour le savoir : cela fait longtemps que je sais où se trouvent ces deux départements. Le droit qui régit

la Moselle, c'est quand même un peu court ! La Moselle, comme le Bas-Rhin, est un département frontalier de l'Allemagne et je ne vois pas comment l'on peut discuter d'une politique transfrontalière de part et d'autre de la frontière franco-allemande si l'on fonctionne de manière distincte.

de cohérence et d'une certaine dignité. Chacun a le droit d'avoir ses idées, mais on ne peut pas dire noir et voter blanc ou bien dire blanc et voter noir. C'est cela qui est insupportable dans notre démocratie. Je voudrais faire une remarque, rejoignant

ce texte pose aussi un problème, celui de graver dans le marbre, si cet amendement n'était pas adopté, une rupture d'égalité entre les départements dans une République que l'on dit une et indivisible.

Un peu dans le même esprit que Jean-Marie Bockel, je dirai que je comprends le souhait des territoires, mais il me semble un peu artificiel d'écrire : « Nous aussi, nous souhaitons avoir les mêmes compétences. » Je vous propose plutôt d'engager une démarche

Maintenant, je me dis que, si l'amendement n° 61 rectifié est adopté, il laissera la possibilité à tous les territoires de choisir les mêmes choses que ce qu'on propose à l'Alsace. Là, la garantie d'une République une et indivisible

mais être une nouvelle fois terre non pas de différenciation, mais d'expérimentation au profit de tous, c'est-à-dire de tous les territoires, comme elle l'a été pour les fonds européens ou le TER. aussi que la France est riche de ses diversités : se sentir Savoyard, Basque, Berrichon, Corse, Alsacien

Finalement, je crois que la différenciation telle qu'elle a été évoquée par Mme la ministre relève de la révision constitutionnelle, qui n'est pas faite. Je pense donc également

On ne sait plus quoi inventer quand on n'a pas d'idée et qu'on a fait un texte creux- je suis parfaitement d'accord avec mon collègue Brisson.

Eh bien, peut-être est-ce parce que vous n'aviez pas entendu le pays gronder que les « gilets jaunes » sont apparus ! Oui, il y a une demande des élus locaux pour plus de décentralisation, pour une France qui pourrait fonctionner un peu plus à la carte

! Réaménager la carte administrative d'un pays est une chose sérieuse, et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts ! Travaillons sur le statut de l'Alsace, mais, de grâce, ne nous mettons pas à tout fiche en l'air

J'entends bien, je l'ai dit précédemment, les préoccupations des uns et des autres. Par exemple, Daniel Gremillet m'a dit : j'ai entendu ce que vous avez dit hier soir.

même si je comprends les préoccupations, je le répète, des uns et des autres. Je fais une incidente pour vous dire que, naturellement- cela a été dit par Guy-Dominique Kennel si le principe de différenciation était déjà inscrit dans la Constitution, nous n'aurions pas besoin de légiférer.

prévoit qu'un département puisse s'attribuer lui-même des compétences. Cette formule est constitutionnellement très discutable. L'attribution de compétences aux collectivités, vous le savez, est une prérogative du législateur.

Cet amendement s'inspire du principe d'adaptation de la législation, tel qu'il existe pour la Corse, mais dans une version plus allégée, en ce qu'il ne prévoit que le seul ajout de la possibilité, pour la Collectivité européenne d'Alsace, de proposer des modifications ou adaptations des dispositions législatives ou réglementaires, comme le prévoit l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales pour chaque région. Quel

il est nécessaire que cette collectivité puisse être consultée à l'occasion des projets et propositions de loi comportant des dispositions lui étant spécifiques. Je ne vois pas pourquoi ce qui est permis à d'autres serait refusé à la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace.

et le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. La notion de compatibilité induit que le schéma est prescriptif, ce qui est en contradiction avec les termes de la déclaration commune du 29 octobre en faveur de la création de la Collectivité européenne d'Alsace.

de la nouvelle collectivité et le schéma régional, mais aussi le schéma de l'eurométropole de Strasbourg. En effet, cette dernière doit, en vertu de la loi Maptam, dans la mesure où elle est frontalière, « élaborer un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées

que le schéma de l'eurométropole soit compatible avec celui de la Collectivité européenne d'Alsace, les départements étant en train de travailler à la stratégie Oberrhein- Rhin supérieur -, qui fixe d'ores et déjà les grandes orientations.

on va finir par faire disparaître totalement le projet de loi. On est en train de faire une réforme pour l'ensemble de la France. Notre collègue Reichardt a très bien soulevé le problème tout à l'heure. Ce qui m'amuse beaucoup dans cette affaire, c'est que,

à modification. Vous ne pouvez pas, en tant que ministre, ne pas respecter les termes d'une loi sur les métropoles qui a été votée dans cette enceinte.

aurait dû être de rétablir l'Alsace comme région de plein exercice. Ça n'a pas été fait.

précédemment. Cet amendement a pour objet d'associer systématiquement le département de la Moselle à l'élaboration du schéma alsacien de coopération transfrontalière. Il s'agit ni plus ni moins, une fois encore,

j'ai déposé cet amendement qui, vous pouvez le constater, est légèrement différent du précédent et présente l'intérêt de me permettre d'avoir un nouveau temps de parole que j'ai à peu près utilisé, monsieur le président.

de manière transpartisane, à avoir auditionné un certain nombre d'acteurs des relations transfrontalières sur notre territoire, notamment des eurodistricts et des centres d'information des consommateurs. en est ressorti de manière très claire que se posait un véritable problème en matière de coopération sanitaire, malgré la publication de l'accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne signé à Weil am Rhein le 22 juillet 2005.

que le schéma de coopération transfrontalière comprendra aussi un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire concernant les établissements de santé.

Gouvernement ? Cet amendement vise à doter la Collectivité européenne d'Alsace d'une compétence en matière de coopération transfrontalière sur le volet sanitaire. Or cette compétence relève directement de l'État à travers l'offre de soins gérée par l'Agence régionale de santé et l'assurance maladie au titre des dépenses induites. par cet amendement s'oppose aux objectifs de l'accord franco-allemand et, de manière plus générale, à ceux des accords transfrontaliers conclus par la France. Les accords de coopération transfrontalière en matière sanitaire, notamment l'accord conclu entre l'Allemagne et la France et signé en 2005, sont des sont des accords-cadres destinés à favoriser la mobilité des patients et des professionnels de santé et à optimiser l'offre de soins dans le cadre d'un diagnostic territorial partagé et adapté aux réalités locales. Sur la base de ces accords-cadres, des conventions locales de coopération sanitaire permettent aux bénéficiaires de l'assurance maladie française et étrangère se trouvant dans les régions frontalières d'avoir accès à des soins de qualité : secours d'urgence, soins programmés, pathologies chroniques. Afin d'avoir une déclinaison au plus près du terrain, les conventions locales de coopération sont négociées et conclues par les acteurs locaux, qui ont une analyse fine de la situation- il s'agit, pour les autorités françaises, de l'Agence régionale de santé Grand Est -, en partenariat avec l'assurance maladie. En l'absence de convention, un patient français a la possibilité de se faire soigner en Allemagne dans le cadre du droit européen. En cas de soins programmés, le patient doit nécessairement obtenir un accord préalable de la CPAM, sans lequel il risquerait de se voir appliquer des tarifs privés et un reste à charge très important. Je me permets d'interpréter votre amendement, monsieur Bigot, comme un amendement d'appel. Il me paraît en effet évident que votre intention n'est pas de donner à la Collectivité européenne d'Alsace compétence en matière de sécurité sociale. Les éventuelles difficultés d'application de l'accord-cadre auront vocation à être examinées par le futur comité de coopération transfrontalière prévu par le nouveau traité d'Aix-la-Chapelle, lorsqu'il sera ratifié.

ministre, que vous nous disiez que cette compétence relève de l'Agence régionale de santé prouve bien que, contrairement à ce qui commence à être annoncé par le Gouvernement, vous n'envisagez pas de véritable décentralisation. La déclaration de Matignon, c'est d'abord le Grand Est qui n'accepte pas, sauf délégation exceptionnelle par convention, de donner une compétence à la Collectivité européenne d'Alsace, qui est un département. Tout à fait ! Par ailleurs, vous laissez entendre que l'État

vote. Je comprends tout à fait la problématique, mais je m'abstiendrai sur cet amendement. Je ne pense pas que le fait d'inscrire dans la loi la compétence sanitaire changera quoi que ce soit sur le territoire.

Or ce sont là des prérogatives de l'éducation nationale et qui doivent le rester. Cet alinéa prévoit aussi l'enseignement immersif. Ce mot pose problème. À strictement parler, l'enseignement immersif est un enseignement exclusivement en langue étrangère ou régionale, contrairement à l'enseignement bilingue, que nous voulons promouvoir. Cet enseignement immersif est possible dans des écoles privées, comme les écoles Diwan, mais pas dans les écoles publiques, car on ne peut pas raisonnablement l'imposer aux parents. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel a jugé qu'un enseignement immersif à l'école publique est inconstitutionnel.

la mise en oeuvre de cet enseignement. De telles dispositions sont déjà prévues dans le cadre de la convention quadripartite. Leur inscription dans le projet de loi a donc plutôt une valeur programmatique.

est à Mme Laurence Harribey. Cet amendement vise à donner la possibilité au président du conseil départemental d'Alsace de recourir à un programme-cadre en matière de coopération transfrontalière régionale.

Un tel mécanisme de simplification existe déjà pour les régions et les départements d'outre-mer. Il a été introduit par la loi de décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération

au traité d'Aix-la-Chapelle, qui a pour objectifs d'éliminer les obstacles dans les territoires frontaliers à la mise en oeuvre de projets transfrontaliers et de faciliter la vie quotidienne des habitants

la commission ? Cet amendement tend à donner à l'Alsace le pouvoir de négocier et de signer, sous certaines conditions, des accords internationaux avec plusieurs États, territoires ou organismes régionaux étrangers. En matière de coopération décentralisée, il est déjà possible pour une collectivité locale française de contractualiser avec des autorités locales étrangères. C'est prévu dans le code général des collectivités territoriales.

vous évoquez, madame la sénatrice, se situent dans la droite ligne de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui invite à tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières des régions ultrapériphériques, et de l'article 73 de la Constitution, qui en tire, dans son premier alinéa, les conséquences pour les départements et régions d'outre-mer dans notre ordonnancement constitutionnel interne. Vous conviendrez conviendrez que ces fondements, tant constitutionnels que géographiques, ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas de la Collectivité européenne d'Alsace. je vous rejoins sur le fait que le dialogue a vocation à se tenir dans le cadre du futur comité de coopération transfrontalière prévu par le traité d'Aix-la-Chapelle. Ce comité sera chargé d'analyser les besoins et de recommander les évolutions jugées nécessaires, y compris, le cas échéant, par un accord international avec la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement ne peut donc

Madame la ministre, avez-vous véritablement pour seul objectif, dans ce projet de loi, de leurrer les Alsaciens ? On insiste sur l'appellation « Collectivité européenne d'Alsace »,

le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre ». Pour quel motif

Cet amendement tend à supprimer le rôle de chef de file de la Collectivité européenne d'Alsace dans la promotion de la langue régionale, introduit par la commission des lois. Une telle suppression s'inscrit dans le droit fil de l'article 104 de la loi NOTRe, qui a fait de la promotion des langues régionales une compétence partagée par tous les échelons de collectivités. Cette compétence partagée permet une diversité des initiatives des collectivités, en fonction des besoins de leur territoire. Dès lors, confier un chef de filât dans ce domaine à une collectivité pourrait contraindre ces initiatives. En outre, la Collectivité européenne d'Alsace pourra, à droit constant, définir un plan de soutien à la langue régionale sans qu'il soit nécessaire de recourir à la loi pour ce faire. Par ailleurs, instituer un chef de file, sans indiquer les conditions concrètes de mise en oeuvre de cette disposition, est source d'incertitudes. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement n'est pas favorable à cet ajout, dont il demande la suppression.

avec les autorités locales étrangères. C'est prévu par le code général des collectivités territoriales. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire. En matière de bilinguisme, la Collectivité européenne recruter et de faire intervenir des enseignants d'allemand pendant les temps complémentaires, c'est-à-dire hors du temps scolaire, organisés par le département. Elle

influe directement, cela a été dit, sur la capacité d'embauche de nos jeunes. Dans certaines communes frontalières, plus de 60 % des actifs travaillent de l'autre côté de la frontière, notamment au Luxembourg ou en Belgique.

Ni l'Alsace, ni la région Grand Est, ni aucune région de France n'ont la compétence en matière d'éducation nationale. Les collectivités locales gèrent les écoles, les collèges et les lycées, mais il s'agit du patrimoine bâti et des équipements de ces établissements.

c'est-à-dire que la collectivité territoriale française ne peut pas, et c'est naturel, s'engager au nom de l'État, qui seul a la compétence éducative. Cette asymétrie dans la coopération est désagréable, dans la coopération est désagréable, mais nous ne pouvons pas, pour régler ce problème de négociations

le Land allemand, qui impose ses exigences sur les programmes scolaires, les qualifications des enseignants, qui est donc tout à fait qualifié pour se prononcer sur les matières éducatives, ait en face de lui une institution dotée des mêmes qualifications, et cela ne peut pas être le cas de l'Alsace, pas plus que de la région Grand Est. Si bien que, mes chers collègues, vous adopterez ou non cet amendement, mais la position de la commission est, elle, très ferme c'est la différence de système entre l'Allemagne et la France qui empêche absolument d'engager, du côté français, l'exercice de la compétence éducative dans un accord transfrontalier. Je ne vois pas comment nous pourrions revenir sur ce point, parce que, demain, ce sont aussi les programmes scolaires, les qualifications requises pour enseigner qui pourront être négociés de part et d'autre du Rhin, du côté français par une collectivité qui n'a pas la compétence et du côté allemand par une collectivité qui l'a. Je ne comprends pas comment on pourrait remettre en cause ce système à la faveur d'une discussion sur le statut de l'Alsace, que nous érigeons en Collectivité européenne d'Alsace. On peut le déplorer, mais c'est une réalité fondamentale dans l'organisation de nos deux pays. La parole est

je tiens à préciser qu'il s'agit d'une carence nationale. L'année dernière, 72 postes ouverts au Capes d'allemand n'ont pas été pourvus

que le chef-lieu de la Collectivité européenne d'Alsace soit situé à Colmar. En premier lieu, le présent amendement entend permettre au préfet de région d'être déchargé du contrôle de la nouvelle collectivité, son activité étant déjà bien lourde par ailleurs. Ainsi, le préfet départemental vérifiera la légalité dans la limite du territoire de la Collectivité européenne d'Alsace et le préfet de région continuera son action sur les territoires de la collectivité Grand Est, en évitant toute confusion entre les deux collectivités. En second lieu, cet amendement entend permettre de conforter la pérennité de la préfecture du Haut-Rhin, qui sera inscrite dans la loi, à l'instar de Strasbourg qui a été désigné chef-lieu de la région Grand Est. La préfecture de Colmar ne pourra ainsi pas être remise en cause par voie administrative. Je tiens à préciser, mes chers collègues, que cet amendement n'implique en rien

que les choses peuvent évoluer. C'est la raison pour laquelle je souhaite sanctuariser le fait que le chef-lieu de la Collectivité européenne d'Alsace soit situé à Colmar.

L'article L. 3621-3 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil départemental. Je pense qu'il faut faire la même chose : « Le chef-lieu de la Collectivité européenne d'Alsace

deux acceptions différentes : c'est la commune dans laquelle est située la préfecture, mais aussi une qualité honorifique reconnue à la principale ville du département.

Pour autant, je suis favorable aux arguments développés à l'instant par notre collègue rapporteur et par la ministre.

M. Loïc Hervé, pour explication de vote. Je profite de l'examen de ces deux amendements pour faire part à nos amis Alsaciens de mon étonnement en découvrant qu'il n'y aurait pas d'adéquation entre le périmètre de la Collectivité européenne d'Alsace et les circonscriptions administratives de l'État. de l'État. Pour avoir assisté à un certain nombre de débats locaux dans le cadre du grand débat national, je vous assure que nos compatriotes ont besoin de lisibilité

administrative de notre pays. La notion même de département en tant que circonscription administrative de l'État, comme de département en tant que collectivité territoriale, qui ne s'appelle pas département mais Collectivité européenne d'Alsace, crée une ambiguïté, et pas seulement pour les Alsaciens, mais aussi pour nos compatriotes. Par ailleurs, le président, l'exécutif de la Collectivité européenne d'Alsace aura pour interlocuteur deux préfets,

totalement disproportionné par rapport à la période significative que nous vivons et qui mérite de la clarté.

beaucoup d'entre vous connaissent certainement des difficultés similaires dans leurs territoires. Vous pouvez donc comprendre qu'il n'est pas forcément utile de créer des problèmes là où il n'y en a pas. La parole est à M.

M. André Reichardt. La politique de formation professionnelle et d'apprentissage présente en Alsace diverses caractéristiques, en ce qu'il subsiste encore une réglementation locale de l'apprentissage et des traditions spécifiques en matière de métiers. Il est en outre reconnu que la formation professionnelle doit tenir compte des possibilités offertes par le marché de l'emploi et des opportunités d'affaires en Suisse et en Allemagne. À cet égard, il est nécessaire de rechercher une meilleure harmonisation des formations et des qualifications avec ces pays. L'enseignement bilingue doit également être renforcé et valorisé dans le domaine de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Partant du constat que de nombreuses difficultés demeurent encore, du fait notamment de la rigidité de règles nationales peu adaptées au contexte local, le présent amendement tend à conférer à la Collectivité

également à prévoir la possibilité pour la Collectivité européenne d'Alsace de signer des conventions avec ces mêmes sociétés pour la diffusion d'émissions en langue régionale, avec des sociétés privées ou des autorités nationales ou étrangères.

Haut-Rhin doit se faire sans qu'il en résulte un éloignement du service public pour les usagers. Sans doute les départements organisent-ils déjà des services déconcentrés territoriaux. Toutefois, il me paraîtrait opportun qu'ils puissent déléguer la mise en oeuvre de l'aide sociale à des collectivités territoriales de niveau inférieur. Cela est déjà prévu pour les métropoles, mais il n'y a pas de raison de limiter cette possibilité à ce dernier type de collectivité dans le cas de l'Alsace. Il convient donc que

il est à préciser que ces actions relèvent certes de l'État et des conseils régionaux, mais avec une possibilité de délégation aux départements qui en font la demande, selon les termes de la loi Maptam.

à l'amendement n° 106 rectifié, qui nous semble satisfait par le droit en vigueur. Les collectivités peuvent d'ores et déjà adresser au Gouvernement des propositions relatives à la promotion des langues

les prestations d'aide sociale, c'est quand même le minimum que l'on doit à nos concitoyens ! La parole

de santé, de mobilité et de formation professionnelle. Comme cela a été dit précédemment sur la question de la langue, la situation de nos voisins est très différente de la nôtre : ils ont un marché de l'emploi très dynamique, une tradition industrielle forte et une démographie extrêmement pénalisante. Quand on examine leurs plans à dix ans, on s'aperçoit qu'ils ont de gros besoins de main-d'oeuvre,

un schéma de formation professionnelle adapté à cette réalité frontalière. Je mets aux voix

de frontières européennes. Au sein de cette Lotharingie, la Haute-Savoie trouve une place tout à fait particulière. Si les Alsaciens ont été précurseurs, il est nécessaire que, dans plusieurs domaines, la coopération transfrontalière puisse être confiée à un interlocuteur C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues de Haute-Savoie Sylviane Noël et Cyril Pellevat, ainsi que Mme Berthet, sénatrice de la Savoie, et d'autres collègues, j'ai déposé cet

qui étend la possibilité à tous les départements de solliciter l'application de l'article 1 du projet de loi. Quel est

l'Agence pour le développement et l'industrialisation de la région Alsace, l'Adira, pourra se voir confier cinq blocs de compétences : le développement économique- 55 % du budget

est chargé d'animer et de coordonner l'action des collectivités et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. Ma question est simple : où est passé le développement économique dans ce texte ? Devant le silence du projet de loi à cet égard, la commission des lois a bien voulu intégrer un de mes amendements visant à rendre cette nouvelle collectivité d'Alsace compétente « pour promouvoir l'attractivité de son territoire en France et à l'étranger Elle n'a cependant pas pu examiner mon amendement n° 89, qui aurait permis à la collectivité d'Alsace de « favoriser l'activité économique sur son territoire par l'organisation et le financement d'organismes de développement ou par des conventions passées avec des organismes existants ». une nouvelle fois, cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances. Je me dois donc de faire ici le même constat que précédemment. Alors que la question essentielle de ce texte est celle des compétences que l'on souhaite attribuer à la Collectivité européenne d'Alsace, le législateur est empêché de débattre à cet égard à cause d'une interprétation de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances. Je ne peux être d'accord avec cela, et je souhaitais le dire explicitement ce

elle doit pouvoir mettre en oeuvre toutes les actions utiles et nécessaires à la valorisation et à la promotion de la destination Alsace, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. Elle doit pouvoir fixer, à l'échelle de l'Alsace, une stratégie globale de développement touristique

laisse pendante la question d'un désengagement futur de l'État de la gestion des grandes infrastructures. De plus, il n'est pas prévu de coordination avec les départements limitrophes et la région Grand Est, alors que les décisions du nouveau département pourraient avoir un fort impact sur les territoires limitrophes. Enfin, après le fiasco de la privatisation des autoroutes, il serait peut-être bon de mieux penser et préparer ce type de transfert. Nous sommes d'ailleurs inquiets des projets de privatisation des réseaux routiers secondaires-